Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance

Même si la loi NOTRe a permis une avancée dans ce domaine, les maires des communes de résidence ne sont pas strictement tenus de participer financièrement. Ils sont invités à à trouver un accord avec les maires des communes d'accueil. À défaut, le préfet peut aussi être sollicité dans l'intérêt de l'enfant, mais il arrive parfois qu'aucun accord ne soit trouvé.

Vous comprendrez que ce n'est pas une décision complètement évidente à mettre en oeuvre et qu'elle ne peut se prendre indépendamment des maires. « C'est pourquoi nous nous sommes mis d'accord, avec Loïg Chesnais-Girard, pour laisser aux communes de Bretagne, représentées au sein de la conférence territoriale de l'action publique, et à la CTAP plus globalement, le soin de se prononcer sur la possibilité d'élargir le forfait scolaire aux écoles bilingues sous contrat.

Longeot. Une reconnaissance plus explicite de l'enseignement bilingue en français et en langue régionale lors des examens ou à l'occasion des thèses et des mémoires permettrait la valorisation des parcours bilingues. Elle aurait également l'avantage de prendre en compte les aspirations des jeunes bilingues passant des examens comme le baccalauréat ou le brevet des collèges. Quel est l'avis de la commission ?

Or la CTAP n'est pas une instance décisionnaire et les petites communes, qui sont les plus concernées par ce dispositif, y sont sous-représentées. Deuxièmement, le forfait scolaire étant, le cas échéant, versé directement par la commune de résidence à l'établissement privé sous contrat, l'accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence n'a pas lieu d'être. sa rédaction est tellement alambiquée que le dispositif de cet article ne constitue pas une obligation de contribuer. Si tel était le cas, cela représenterait une charge considérable pour les communes, particulièrement les plus petites, qui ne ferait l'objet d'aucune compensation. L'article 6 A devra faire l'objet d'une réécriture. C'est pourquoi je regrette l'absence d'initiative du Gouvernement. S'agissant de la transcription d'un engagement pris par lui, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement sur les amendements n 389

Toutefois, il n'est pas opportun de les placer en position d'autorité à l'égard des enseignants, et encore moins de les faire participer à leur évaluation aux côtés des inspecteurs de l'éducation nationale, d'autant que les consultations avec les syndicats ne sont pas encore terminées.

Il introduit une disposition lourde de conséquences pour les enseignants, sans avoir fait l'objet d'aucune concertation avec les personnels concernés. Ainsi, au détour de l'adoption d'un amendement, les « maîtres d'école », pour reprendre l'appellation maintenue dans l'article L. 411-1 du code de l'éducation, vont se retrouver placés sous l'autorité du directeur d'école, qui, de surcroît, participera à leur évaluation, en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale- une formulation par

débattons-en ! Creusons la question, mais nous ne la réglerons pas simplement en créant un lien hiérarchique entre le directeur et l'équipe enseignante. Qui plus est,

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande

Le scrutin est ouvert.

Mme Marie-Pierre Monier. Notre amendement vise à maintenir le rôle de simple coordination du directeur d'école entre les maîtres et à l'étendre aux autres personnels de l'école. Nous proposons de compléter le dispositif afin de prévoir une concertation entre le directeur et la commune pour l'organisation des activités périscolaires.

Le scrutin est ouvert.

je vais donner lecture d'un passage de l'article L. 411-1 du code de l'éducation, qui précise le rôle du directeur d'école maternelle ou élémentaire : « Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres

C'est important pour la réussite et l'épanouissement de tous les élèves. Les directeurs d'école assument toutes les responsabilités, ils sont les interlocuteurs de leur propre autorité hiérarchique, hiérarchique, des enseignants, de l'équipe éducative, de la mairie, des enfants, des parents. Bref, ils sont les « couteaux suisses » de l'école de la République et, ne serait-ce qu'à ce titre, ils mériteraient que la question de leur statut soit réglée définitivement.

et l'administration, d'autre part, sur l'ensemble des questions relatives à la vie scolaire. Ce sont le plus souvent des retraités, fréquemment d'anciens personnels de l'éducation nationale. Leur mission, initialement circonscrite

Nous comprenons les inquiétudes qu'a suscitées cet article : il s'agit d'une disposition importante, introduite sans avoir fait l'objet d'une étude d'impact. De plus, ce projet n'a pas fait l'objet de concertations suffisantes. Cependant, loin de signer l'arrêt de mort des écoles ou des directeurs, la mise en oeuvre de ce dispositif permettrait de créer un vrai continuum entre le primaire et le collège, au bénéfice des élèves. Il convient donc de rétablir l'article dans une nouvelle rédaction, plus précise, en y intégrant certains gages de sécurité, comme la consultation des conseils de l'école et du conseil d'administration du collège, sachant que ce nouveau dispositif n'a pas vocation à être obligatoire. Il convient de donner toutes les chances à nos enfants et de leur offrir une école véritablement inclusive. Quel

Or le Sénat est la voix des élus. Que ces inquiétudes, ces crispations n'aient pas toujours reposé sur une lecture attentive du texte, je peux en convenir, mais nous

fixe un objectif. Elle pose que le dispositif est un outil d'aménagement éducatif à la main des élus locaux, en particulier de ceux qui sont confrontés à la déprise démographique de leur territoire.

d'une part, le secteur du collège, auquel il est fait référence, demeure déterminé par le seul conseil départemental ; d'autre part, la participation ou non des écoles relève de la seule décision des collectivités volontaires.

Ce grand principe pédagogique et éducatif s'accompagne d'un certain nombre d'autres considérations. La première d'entre elles, c'est que l'on observe des formes de décrochage en classe de sixième parce que le continuum entre

des enjeux actuels, entre la commune et l'école. À la lumière de ces inquiétudes, certains de nos collègues ont jugé bon de retravailler

Or, au sujet des établissements publics des savoirs fondamentaux, leur réponse est sans appel. Certes, il s'agirait de regroupements facultatifs, menés sur l'initiative des collectivités territoriales, mais de nombreux maires m'ont fait part de leur légitime inquiétude.

les services publics sont en régression permanente : toujours moins de services publics, toujours moins de bureaux de poste, toujours moins de services de santé ! Allons-nous maintenant organiser la suppression de classes et d'écoles,

pour le temps long. C'est se laisser traverser par tout ce que le pays murmure. C'est ne pas se contenter d'une vision comptable, à court terme. En définitive, que voulons-nous pour notre pays ?

nous allons en rester à la suppression de l'article 6 Je remercie néanmoins Jacques Grosperrin du patient travail qu'il a mené pour tenter de trouver une solution de compromis. Ce travail ne sera pas inutile, car il contribuera à la poursuite du débat dans les semaines et les mois qui viennent.

: notre objectif est au contraire de renforcer l'école primaire au cours des prochaines années. Non, il n'y aura pas de remise en cause de la fonction de directeur d'école, ni de diminution du nombre de directeurs d'école ; je suis le premier à penser qu'ils sont extrêmement utiles, que leur fonction est fondamentale et que nous avons besoin de les renforcer. Sur ces trois sujets,

la délibération du conseil municipal sur les mesures de retrait ou de maintien de postes au moment de l'élaboration de la carte scolaire. Nous pensons, monsieur le ministre, que cette mesure serait de nature à redonner du crédit

Le scrutin est ouvert.